je ne porterai pas la loi NOTRe comme une croix. Cette loi n'était pas parfaite- tant s'en faut ! Nous le savons maintenant et nous nous devons de le reconnaître, afin de prendre les mesures qui sont nécessaires pour en corriger les effets négatifs.

est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Pierre Grand. Sur le modèle des dispositions récemment entrées en vigueur pour la création de communes nouvelles, il paraît important que toute décision de modification d'un périmètre soit accompagnée d'éléments financiers permettant aux élus d'en appréhender au mieux les conséquences. Il convient également que les citoyens soient informés de ces éléments. Je propose donc de prévoir la mise en ligne sur internet du document présentant les incidences financières de la modification du périmètre de l'EPCI.

Nous proposons très simplement de procéder à l'élection du maire et des adjoints de façon concomitante par scrutin de liste à la majorité absolue. C'est une manière non seulement de témoigner de la solidarité de l'équipe municipale, mais surtout de garantir une parité réelle,

Il faut rappeler qu'on dénombre seulement 17 % de femmes parmi les maires, et 29 % parmi les premiers adjoints. C'est encore beaucoup trop faible. Deux raisons à cela. D'abord, il n'y a pas de scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants, à la fois pour l'élection des conseillers municipaux et pour celle des adjoints. Ensuite, et surtout, si les listes alternatives homme-femme ou femme-homme sont obligatoires pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants, s'agissant de la liste pour les fonctions d'adjoint, la loi impose seulement que l'écart entre le nombre de candidats ne soit pas supérieur à un. Elle n'exige donc pas une alternance stricte femme-homme dans la liste de candidats. Nous souhaitons par conséquent imposer au moins la parité au sein du binôme constitué par le maire et son premier adjoint, afin de favoriser la féminisation des exécutifs communaux, ce qui aura également pour conséquence de féminiser les conseils communautaires. Je vous remercie

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses lois ont permis de faire considérablement progresser la parité en politique. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, l'AMF, ainsi que l'Association des maires ruraux de France, l'AMRF, et plusieurs autres associations d'élus locaux ont cependant souligné, à juste titre, que des progrès restaient à faire dans certains domaines, notamment au sein des exécutifs des collectivités territoriales. L'Association des maires ruraux de France a, par exemple, réclamé à plusieurs reprises la suppression du seuil de 1 000 habitants, afin que le scrutin de liste avec obligation de parité soit étendu à toutes les communes. L'AMF et l'AMRF ont également suggéré que, dans les municipalités, le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Enfin, une demande encore plus insistante a été formulée pour que l'obligation de parité s'applique aux vice-présidents des intercommunalités sur la même base qu'aux adjoints dans les communes. Malheureusement, malgré cette convergence d'avis, le Gouvernement semble ne pas considérer que cette problématique soit prioritaire.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les règles de parité appliquées aux adjoints au maire présentent deux lacunes. Tout d'abord, la parité se limite aux adjoints et ne prend pas en compte le maire. De ce fait, une commune, par exemple de 1 200 habitants, qui a trois adjoints, a souvent un maire et deux adjoints de même sexe, ce qui conduit à un ratio de parité fort peu satisfaisant. Par ailleurs, en cas d'élection partielle à des postes d'adjoint, la jurisprudence exige que la parité s'applique séparément aux sièges à pourvoir. Si, par exemple, quatre femmes adjointes au maire ont démissionné, la municipalité est obligée d'élire non pas quatre nouvelles adjointes, mais deux adjointes et deux adjoints.

Il faut cependant rappeler que nous sommes tenus par des exigences politiques et constitutionnelles, que nous ne pouvons pas ignorer dans cette maison. Aussi, nous proposerons d'aller le plus loin possible

que le premier adjoint soit de sexe différent que le maire. Le Sénat a déjà examiné cette proposition deux fois, en 2014 et 2016,

collègues proposent, comme une avancée, qu'elle soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. C'est ce que l'on appelle communément la « liste chabada ». Cela ne bouleverse pas du tout le fonctionnement du conseil municipal.

C'est donc de la pédagogie de répétition ! Il n'en demeure pas moins que vous confondez le moyen et la finalité. En l'espèce, qu'est-ce que le fait qu'il y ait une élection de liste et que le maire soit le premier va changer ? On sait que le premier ou la première aura toute la latitude et les prérogatives du maire. C'est clairement identifié, et cela ne pose aucune difficulté, mais il est toujours facile d'invoquer la tradition quand on ne veut pas avancer. Par ailleurs, je vous rappelle qu'en France le maire est déjà

non pas au fait d'être premier, deuxième, troisième ou quatrième adjoint, mais à une répartition assez sexuée des compétences et des attentes des uns et des autres dans une vision genrée des responsabilités électives, même si, Annie Guillemot l'a rappelé la semaine dernière, ce constat

Durain, la tradition n'est pas le sujet. Quand on dit que le maire est élu traditionnellement, cela ne veut pas dire que l'on est traditionaliste. Cela signifie que le maire, par ce qu'il incarne,

distinguent bien des autres. C'est important à mes yeux. J'ai bien expliqué que, juridiquement, on ne peut pas lier deux élections. Pour terminer, je ne voudrais pas laisser croire que la commission des lois

à M. le ministre. Monsieur le sénateur Kerrouche, le parallèle avec les conseils départementaux et les conseils régionaux ne peut pas être fait puisque vous avez un droit et une pratique dans les collectivités départementales et régionales.

Je le dis une fois de plus, madame la rapporteure, je ne trouve pas que la modification du mode de scrutin pour les vice-présidents d'intercommunalité soit forcément ce que nous avons fait de mieux la semaine dernière. Vous connaissez mes opinions sur le sujet. Je vous propose de ne pas modifier désormais l'ambiance et la gouvernance au sein des communes.

Cela peut poser problème, notamment lorsqu'un adjoint se voit retirer ses délégations tout en étant maintenu en fonctions par le conseil municipal. Dans ce cas-là, le maire est obligé de lui redonner une délégation, même minime. Sinon, il ne peut pas accorder de délégation à des conseillers ; il doit même retirer les délégations qu'il a pu confier préalablement à des conseillers municipaux. Mon amendement vise à supprimer cette restriction pour faire en sorte que le maire puisse librement accorder des délégations aux conseillers municipaux, municipaux, sans qu'il y ait d'incidence sur l'enveloppe des indemnités, quelle que soit la situation des adjoints, qu'ils aient ou non tous une délégation. Quel est l'avis de la commission ? Le président

est, en soi, extrêmement saine : un maire ne peut déléguer une partie des attributions à de simples conseillers municipaux que si tous les adjoints sont pourvus de délégation.

me semble un peu étrange par rapport à la définition d'origine de la loi. Toutefois, je conviens qu'on est parfois confronté à de telles situations,

Or il est de moins en moins exceptionnel qu'un maire modifie son exécutif en cours de mandat en retirant des délégations à un ou plusieurs adjoints, appelant ainsi le conseil municipal à se prononcer sur leur maintien ou non. Si cette faculté a été mise en place pour éviter des blocages, certains maires ou présidents d'intercommunalité peuvent s'en servir afin de mettre la pression sur certains adjoints ou vice-présidents et ainsi modifier leur exécutif au gré des humeurs. Dès ses premiers arrêts en la matière, le Conseil d'État exigeait que le motif du retrait des délégations de l'adjoint ne soit pas étranger à la bonne marche de l'administration municipale, concept très large, puisque toute tension au sein de l'équipe communale peut entrer dans ce cadre. L'amendement n° 38 vise donc à mieux encadrer ces retraits par la mise en place d'un scrutin secret- après tout, c'est le parallélisme des formes -pour la décision de maintien ou non d'un adjoint et par une limitation des possibilités de retrait au risque d'appeler le conseil municipal à se prononcer sur le maintien ou non du maire dans ses fonctions.

la remise en cause du mandat du maire. Le Conseil d'État l'a rappelé à plusieurs reprises, le maire est le seul chef de l'administration communale. Le droit en vigueur me semble suffisamment équilibré pour perdurer en l'état. Vous proposez une élection à bulletin secret quand le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien en fonctions d'un adjoint.

Moi, je suis responsable devant vous, et encore plus devant l'Assemblée nationale, selon les termes de la Constitution. Le maire n'est pas responsable devant son conseil municipal. D'ailleurs, quand il n'a pas de majorité, il ne tombe pas pour autant. Il faut vraiment des circonstances très particulières pour que l'État reprenne la main sur une collectivité qui ne fonctionnerait plus du tout.

L'élection d'un adjoint ou d'un vice-président se fait à scrutin secret. Je pense qu'il est plus cohérent de prévoir que

par un scrutin de liste paritaire, le premier vice-président soit de sexe différent du président. Rappelons-le en effet, la loi prévoit que les exécutifs départementaux et régionaux sont paritaires. La parité est atteinte pour les postes de vice-président, qui sont occupés à 48,4 % par des femmes. En revanche, les femmes n'occupent les postes de président respectivement que dans 9,9 % et 16,7 % des cas. Les postes de premier vice-président ne sont dévolus à des femmes que dans 34,7 % des cas dans les départements et dans 27,8 % des cas dans les régions, alors que ce sont des assemblées paritaires ! Cet amendement vise à remédier aux inégalités qui subsistent entre femmes et hommes au sein des exécutifs locaux et prévoit que les titulaires des fonctions de président et de premier vice-président sont nécessairement de sexe différent. Cette disposition, qui s'applique aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, ainsi qu'à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse, à la

je veux parler du vrai pouvoir. La présence des femmes en bonne place dans les exécutifs est plus que jamais nécessaire dans un souci de simple respect des uns et des autres, en l'occurrence des femmes, afin qu'elles aient leur place, toute leur place. C'est une question de justice, en somme ! La parole

Merci,

aux inégalités qui subsistent entre femmes et hommes au sein des exécutifs locaux. Ces mesures sont réclamées de longue date par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, et également proposées par l'AMF, les associations de femmes élues et les associations nationales d'élus locaux. Peu à peu, nous constatons une convergence transpartisane sur l'urgence à trouver des solutions pour faire avancer la parité dans les lieux de pouvoir local. Les modalités proposées par les uns et les autres peuvent varier, mais l'objectif est identique : la parité dans les conseils et les exécutifs des collectivités locales. Cet amendement, s'il est adopté, serait un grand pas en avant pour la visibilité des femmes en politique et pour un réel partage du pouvoir dans nos territoires. La parité, rappelons-le, est une exigence de justice et de démocratie. Et selon Mme Danielle Bousquet, ancienne présidente du HCE, compter sur la bonne volonté et l'histoire est une douce utopie dans ce domaine. Nous le savons, c'est avec l'adoption de contraintes légales que la parité progresse au sein de la majeure partie des assemblées locales et des bureaux. À défaut, les fonctions exécutives locales restent largement l'apanage des hommes. Lorsque des contraintes paritaires sont appliquées, le partage du pouvoir est une réalité. Quand la parité est aujourd'hui effective dans les assemblées délibérantes, elle ne se traduit que rarement dans les exécutifs locaux. La parité est en trompe-l'oeil : les femmes n'occupent les postes de présidente de conseil départemental que dans 9,9 % des cas et elles ne sont que 16 16 % des maires sont des femmes. Oui, la nouvelle étape de la parité, c'est bien la parité dans les exécutifs locaux, notamment pour les fonctions de présidente et de vice-présidente. C'est le nouveau plafond de verre qu'il nous faut briser. C'est par la loi que nous permettrons de casser cette forme d'autocensure que peuvent connaître les femmes dans les territoires. Le moment est

Cela reviendrait à dire, si je comprends bien, qu'on peut contourner la difficulté dont nous parle Mme la

qui visait à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires. Ce texte a été adopté à une large majorité par le Sénat. Le présent amendement vise à modifier les règles relatives à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre, afin d'assurer une plus juste représentation des communes de taille moyenne. Selon les règles actuelles, chaque commune est bien représentée au sein de ces assemblées. Mais les communes dont la population se situe autour de la moyenne communautaire sont pénalisées.

reprend l'article 1 d'une proposition de loi, qui a été adoptée par la commission des lois du Sénat le 16 janvier 2019 et par le Sénat le 24 janvier

dont se plaignent les élus des petites et moyennes communes, et nous sommes leurs représentants ... Il faut aller dans le sens de l'équité, pour donner plus de place à l'accord

et très contrariant- il est même plus qu'irritant -de la composition des conseils communautaires, c'est-à-dire de la représentation de chacune des communes au sein de ces organes. La semaine dernière, nous avons adopté un amendement, sur proposition de la commission des lois,

de représentation entre communes par rapport à la proportionnelle démographique. Or je vous rappelle, mes chers collègues, que la démographie est le critère essentiel, prioritaire, voire quasi unique, retenu depuis l'arrêt.

pour éviter tout risque de déstabilisation des conseils communautaires qui s'en seraient inspirés pour organiser la représentation de leurs communes. Même si je n'ignore

l'application de votre proposition aux élections de 2026, puisque les organisations de représentation des communes au sein des conseils communautaires ont dû être achevées pour le 31 août.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'étais pas très enthousiaste sur le scrutin de liste dans les intercommunalités : on écarte progressivement les maires ruraux de l'exécutif intercommunal

décision et se demande ce qu'elle fait encore dans cette communauté de communes, avec le peu de représentativité qu'elle y a. Je me félicite de

Pour cette raison, je voterai ces amendements. Il est évident que les petites communes sont spoliées dans le dispositif actuel.

elle n'est pas sortie de nulle part. Deuxièmement, le président du Sénat nomme trois de ses membres. Troisièmement, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui, dans notre pays, est le Constituant. Le Constituant est, soit le peuple français, soit les parlementaires, qui représentent le peuple français. On ne peut pas présenter, notamment aux personnes qui suivent nos débats,

la semaine dernière s'y conforme, et elle permet déjà de résoudre une grande partie du problème. À présent, si nous voulons réellement dégager la voie pour une meilleure représentation des communes dans les intercommunalités, la seule solution

une disposition permettant de revenir sur ce que nous considérons comme des excès de la jurisprudence constitutionnelle, quant à la composition des conseils communautaires.

libellé : La parole est à M. Jean Louis Masson. De 2007 à 2017, les présidents Sarkozy et Hollande ont voulu réorganiser l'administration territoriale autour de structures administratives démesurément étendues.

Toutefois, cette problématique est encore considérablement aggravée par les fusions arbitraires ayant conduit à des régions et à des intercommunalités tellement grandes qu'il n'y a plus aucune gestion de proximité.

On aurait pu admettre que les deux départements alsaciens ou les quatre départements lorrains soient absorbés par les régions d'Alsace ou de Lorraine. En revanche, une opération de ce type à l'échelle de la région Grand Est serait totalement irresponsable. De même, une succession de fusions contraintes à l'échelon des intercommunalités a créé des structures hors sol complètement déconnectées du terrain. Pis encore, les fusions ont presque toujours été faites en bloc, sans découpage pour redistribuer à bon escient le territoire des intercommunalités concernées.

que 303 communes soient situées à plus d'une heure et demie de route du siège de leur intercommunalité ; que 1 766 communes soient à plus d'une heure de ce point et que 7 701 autres soient à plus d'une demi-heure. C'est aberrant Certes, en théorie, une commune peut toujours solliciter un changement d'intercommunalité. Toutefois, les conditions requises sont extrêmement contraignantes, d'autant que le préfet possède ensuite un quasi-pouvoir de blocage. avec cet amendement, nous proposons que toute commune située à plus de trente minutes du siège de son intercommunalité puisse obtenir de plein droit son rattachement à une intercommunalité plus propre,

la parité. Depuis 2013, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'élection des conseillers municipaux se déroule au scrutin proportionnel de liste à deux tours, avec une prime majoritaire et l'application des règles de parité.

dans toutes les communes comptant 1 000 habitants et plus. Pourtant, seuls 16 % des maires et 8 % des présidents d'intercommunalité sont des femmes. Nous devons donc aller plus loin, tout en gardant à l'esprit la réalité du terrain : celle des petites communes et des territoires ruraux, qui font face à une véritable crise des vocations.

Accroître le nombre des communes qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste à la proportionnelle permettra de favoriser la parité et le pluralisme. Nous l'avions déjà proposé en 2013, lors de l'examen de la loi relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux. de janvier dernier, la part des femmes dans les conseils municipaux était de 39 %, toutes tailles de communes et toutes fonctions confondues. Seulement, si l'on regarde les communes de moins de 1 000 habitants, où les candidats sont élus au scrutin majoritaire, donc sans obligation de parité, cette proportion descend à 34 % ; or, dans les communes de plus de 1 000 habitants, elle s'élève à 46,8 %., plus on s'éloigne de fonctions exécutives, plus le nombre de femmes augmente. Le ministère de la cohésion des territoires

de trois mois d'un scrutin. Je le déconseille très fortement, tout en m'en remettant, bien entendu, au vote du Sénat. J'ai demandé un scrutin public pour que chacun prenne ses responsabilités, car je considère que, si nous décidions de changer le mode de scrutin d'un tiers des communes de France au mois de janvier prochain,

quand l'Association des maires de France, l'Association des communautés de France, l'Association des petites villes de France, Villes de France et France urbaine ont signé un texte commun sur la parité, invitant le législateur à prendre des dispositions en la matière le plus rapidement possible.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

en fin de liste soient susceptibles de « monter » en cas de disparition du maire pour permettre que le conseil soit au complet sans provoquer une autre élection.

permettent à une équipe de diriger, mais on peut aussi imaginer que quelques personnes qui n'arrivent pas à composer une liste complète

Le scrutin est clos. Personne ne demande plus à voter ? ... Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater les résultats du scrutin.

n° 202 rectifié . Le ministère de l'intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est déterminée en fonction d'une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pis encore, il n'y a pas de possibilité d'être non-inscrit ou sans étiquette. Conformément au principe de liberté d'opinion de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier, ou à ou à tout le moins, de ne pas se voir attribuer arbitrairement une nuance politique.

L'amendement du président Maurey a pour objet de préciser que dans les communes de moins de 3 500 habitants, l'administration appose une nuance politique uniquement aux candidats ayant choisi une étiquette. Cet amendement a été rectifié,

J'ai bien compris que, pour que la loi ne soit pas bavarde, mes collègues étaient invités à retirer leurs amendements, et que, par instruction aux préfets, jusqu'à 3 500 habitants, on ne demanderait pas, sauf volonté expresse des têtes de liste, l'indication de leur appartenance politique.

lui tout seul. Ainsi, si le maire d'une ville de 8 000 habitants souhaite être sans étiquette et en fait la demande expresse, je ne vois pas pourquoi on lui opposerait un refus et on le mettrait dans une case quelconque. La

au sein ou à la tête d'un syndicat d'un EPCI sans fiscalité propre, alors que la loi NOTRe de 2015 prévoyait que cela ne soit plus possible à compter du 1 mars 2020. Si nous comprenons la volonté d'élargir la représentation des EPCI sans fiscalité propre pour siéger au sein des syndicats mixtes, il n'est pas souhaitable que des personnes non élues accèdent à de telles fonctions. Le comité syndical est l'instance plénière où les décisions importantes sont prises et définit les politiques de gestion et de fonctionnement de l'EPCI. À notre sens, seules des personnes choisies par les administrés et, donc, élues doivent pouvoir accéder Nous proposons par conséquent de supprimer cette disposition et encourageons les citoyens qualifiés à s'engager dans la vie de leur commune comme préalable. Quel

parce que je considère que la démocratie représentative passe par les élus. Le fait de permettre à des citoyens non élus de représenter

permettrait de répondre en grande partie à la préoccupation de ces élus qui se sentent aujourd'hui capables de gérer eux-mêmes la présidence de leur syndicat sans faire appel à des personnalités extérieures.

que la question se pose pour des petites communes rencontrant parfois une difficulté pour se faire représenter dans des syndicats.

À l'évidence, il ne peut être question d'imposer la désignation de représentants des communes en dehors du conseil municipal. Néanmoins, la faculté de le faire peut être précieuse. Je vous citerai un exemple du bocage, mes chers

Le président du syndicat d'eau, qui était le maire d'une commune, âgé de 72 ans, décide de se retirer du conseil municipal. Heureusement, le premier vice-président peut lui succéder à la présidence du syndicat

Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre en place des cellules de reclassement pour anciens élus. Tout à fait ! Je vous le dis comme je le pense, monsieur le président

mais de la fonction si, à force d'accepter de petites dérogations, nous autorisons des gens qui ne sont plus ou pas élus à assurer certaines fonctions ? Personnellement, je pense qu'il faut être élu

du CGCT le même alinéa que celui qui existe déjà à l'article L. 5711-1 applicable aux syndicats mixtes fermés, afin de permettre à un EPCI à fiscalité propre de continuer à choisir, pour l'élection des délégués appelés à siéger au comité du syndicat mixte ouvert dont il fait partie, des membres de son organe délibérant ou bien des conseillers municipaux de ses communes

fiscalité propre, une différence entre les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts. Ainsi, pour l'élection des délégués au comité d'un syndicat mixte fermé, l'article L. 5711-1 du CGCT maintient bien la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de choisir un membre de leur organe délibérant ou tout conseiller municipal d'une commune membre de cet EPCI. En revanche, pour les syndicats mixtes ouverts, les délégués des EPCI à fiscalité propre devront obligatoirement être choisis parmi les membres de leur organe délibérant. Cette différence aura en pratique deux conséquences. D'une part, elle contribuera automatiquement à accroître la charge de travail des seuls élus communautaires ou métropolitains, qui ne sont pas toujours très nombreux. D'autre part, elle aura pour effet de dessaisir de leurs responsabilités un nombre important de conseillers municipaux et de conseillères municipales,

en général, lorsque l'un d'eux siège dans une instance déléguée, il représente d'abord l'instance, en partage et en épouse les ambitions en oubliant parfois l'institution qui l'a mandaté.

de dire que la légitimité des élus est remise en cause, puisqu'en réalité les élus sont appelés dans différentes institutions, mais ils passent leur temps en réunion

l'on peut mettre à la disposition d'un syndicat, sans pour autant trahir le conseil municipal. Enfin, ne pas être élu ne signifie pas que l'on n'a pas la capacité d'assumer un certain nombre de responsabilités

Cette structure a pour mission principale d'évaluer, selon une méthodologie fixée par la loi, les charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique. L'organisation et la composition de cette commission sont précisées de manière succincte par le législateur. Il paraît nécessaire que les préconisations de cette commission ne soient pas remises en cause par des votes en conseil communautaire, dont la composition est très déséquilibrée. cette commission n'intervient qu'une fois les transferts de compétences actés. Or il pourrait être utile d'avoir un aperçu en amont des impacts d'un transfert de compétences en termes de charges transférées. Cet amendement tend à fortifier le rôle de cette commission, en introduisant un volet prospectif dans ses missions.

laquelle a pour mission principale d'évaluer, selon une méthodologie fixée par la loi, les charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique, la FPU. Or cette commission n'intervient actuellement qu'une fois les transferts de compétences actés, remettant dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de compétences un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Je suis convaincu qu'il serait utile pour un EPCI et pour ses communes membres d'avoir un aperçu en amont des impacts d'un transfert de compétences en termes de charges transférées. C'est pourquoi je propose que cette commission,

de révision du montant initialement fixé des attributions de compensation. En dehors de ces procédures strictement limitées de révision unilatérale et de l'hypothèse d'un transfert de charges, il n'est pas possible de prévoir la révision des attributions de compensation sans l'accord des communes concernées, et ce alors même que le montant des attributions de compensation se fonderait sur des éléments erronés ou encore sur des accords financiers devenus caducs. Aucune procédure prévue ne permet donc à l'EPCI de modifier unilatéralement les attributions de compensation et ce dernier peut donc se retrouver contraint de verser des sommes alors qu'il ne perçoit plus par ailleurs En outre, les changements de mandature peuvent également révéler des erreurs dans le calcul du montant de l'attribution de compensation. Or aucune procédure ne permet ni aux communes concernées ni à l'EPCI de procéder à une révision des attributions de compensation pour prendre en compte et rectifier de telles erreurs.

unilatéralement les attributions de compensation, lorsque des versements antérieurs qui relevaient non de transferts de charges, mais d'un accord financier entre l'EPCI et une de ses communes membres ont été intégrés par erreur dans ce flux financier. Quel

professionnelle unique à ses communes membres, pour la raison que le montant des produits fiscaux qu'il perçoit en lieu et place des communes est plus élevé que le coût des compétences qui lui ont été transférées. Voilà pour le principe. Ces Ces attributions de compensation n'ont pas vocation, compte tenu de la définition que je viens de donner, à compenser des versements qui interviendraient dans l'autre sens, c'est-à-dire des communes vers l'EPCI. Leur montant est fixé, soit dans les conditions de droit commun, soit librement par des délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux. L'attribution de compensation due à une commune ne peut être révisée à la baisse qu'avec son accord, sauf en cas de diminution des bases imposables. cet amendement a pour objet d'autoriser une révision unilatérale des attributions de compensation par l'EPCI en cas de diminution ou de disparition d'une somme intégrée dans l'attribution de compensation, indépendamment du strict calcul que j'ai évoqué. Or, en droit, une telle somme ne peut pas être intégrée au calcul de l'attribution de compensation. Votre amendement soulève une vraie question, mais qui est beaucoup plus générale plus générale : dans quelles circonstances est-il opportun de pouvoir imposer à une commune une révision à la baisse de son attribution de compensation Il est vrai que, parfois, les attributions de compensation dans certains territoires ont été calculées un peu rapidement, notamment à la suite des changements de périmètre ou de transferts de compétences qui ont lieu ces dernières années. Il me semble que cette question

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les commissions départementales de la coopération intercommunale sont composées, en ce qui concerne le bloc communal, à 40 % de représentants des communes et à 40 % de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Elles ont ainsi pu constituer un réel contre-pouvoir au préfet, comme en témoignent leurs travaux dans de nombreux départements à l'occasion de l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale de 2011 à 2012, puis en 2016.

des CDCI en diminuant la part des représentants des EPCI à fiscalité propre à 30 % pour augmenter la part des représentants des communes à 50 %. Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à conserver la composition actuelle de la CDCI.

Jusqu'à la loi de décembre 2010, la CDCI était composée de la manière suivante : 60 % de représentants des communes, 20 % de

des représentants des communes ayant baissé à 40 %, avec une petite évolution pour les départements et les régions. S'appuyant sur le principe que les EPCI, donc l'intercommunalité, procèdent de la commune, a jugé nécessaire de modifier cette composition qui avait, en quelque sorte, augmenté la représentation des intercommunalités et baissé celle des communes, en proposant la représentation suivante : 50 % aux communes et 30 % aux EPCI.

car ces collèges sont réservés aux plus grosses communes du département, à celles dont la population est inférieure à la moyenne départementale, à celles dont la population est supérieure à la moyenne départementale, aux syndicats mixtes

Selon les cas, les budgets des conseils départementaux peuvent connaître des déséquilibres, notamment au bénéfice des départements les plus riches. Ce serait inhiber les départements que de passer outre leur accord dès lors que la création d'une commune nouvelle touche des communes issues de départements différents. s'il ressort de la note de cadrage de la commission que les amendements visant à modifier notamment les limites administratives des régions n'ont pas de lien avec le texte déposé, il semble que, par cohérence, il devrait en être de même pour ceux qui tendent à permettre En effet, des communes nouvelles peuvent être créées entre des départements situés sur des limites régionales.

L'Assemblée nationale, pour sa part, n'a pas du tout suivi le Sénat, considérant qu'il appartenait aux acteurs locaux de se mettre d'accord.

Considérant qu'il était difficile pour le législateur de se saisir de ces situations, la commission des lois a proposé que, en cas de désaccord des conseils départementaux, le différend soit tranché par décret.

Est-ce que, nuitamment parfois, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent, par voie d'amendement, modifier le périmètre d'un département

hors sol par rapport à la situation sur le terrain. Je pense que le dispositif tel qu'il est proposé aujourd'hui par la commission va dans le bon sens et qu'il permettra de trouver et